L'attractivité des établissements français, qui a déjà subi les conséquences de l'augmentation des frais universitaires pour les étrangers- nous en avions longuement débattu dans cet hémicycle -, va une fois de plus en pâtir. Ainsi, Campus France va devoir redoubler d'efforts pour attirer et accueillir les étudiants étrangers et aura besoin, pour ce faire, de moyens supplémentaires. Les besoins exprimés s'élèvent, à ce stade, à 3 millions d'euros. Cet amendement vise donc à alimenter l'action n° 4, Enseignement supérieur et recherche

de l'étranger, en particulier de l'association Aledas de Barcelone qui mobilise l'ensemble du réseau de l'AEFE sur la question de l'école inclusive.

Cet amendement de M. Montaugé tend à créer un programme intitulé « Aides d'urgence aux filières agricoles en difficulté à la suite du confinement dû à l'épidémie de covid-19 », alimenté à hauteur de 150 millions d'euros, afin de compenser les pertes de production des agriculteurs durant le confinement.

Lorsqu'un représentant du Gouvernement, quels que soient les sentiments que vous avez envers lui, indique au banc, devant le Parlement, que la France a notifié à la Commission européenne le relèvement des crédits nationaux d'un programme, je pense que cela vaut engagement, et que cela mérite sinon la confiance, du moins le respect des institutions.

par l'ensemble des acteurs d'un même territoire. Ils ont ainsi pour effet de faire émerger des projets répondant à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Ils permettent de favoriser et d'accélérer les circuits courts et intègrent totalement la nécessité de tendre vers l'alimentation locale et de qualité que nos concitoyens appellent de leurs voeux. Cette dynamique est vertueuse à plus d'un titre : elle est bonne pour nos producteurs agricoles locaux, elle est bonne pour les citoyens, puisque

ces dernières années par des politiques injustes et inefficaces alors que, de l'aveu même de la Cour des comptes, ces aides sont un puissant outil de redistribution sociale. La baisse de 5 euros, conjuguée à la non-revalorisation, a conduit ce gouvernement à faire une économie substantielle- on peut

Le rapport de la commission des affaires économiques avait évalué financièrement ces mesures : la suppression du mois de carence coûterait entre 240 et 260 millions d'euros ; la réindexation équivaudrait à 171 millions d'euros.

est ainsi libellé : La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian. Depuis le début du quinquennat, mon groupe demande au Gouvernement une réorientation d'urgence de la politique du logement. Le logement social et le soutien des ménages modestes doivent être au coeur du plan de relance pour la construction et la rénovation. L'État est garant du droit au logement, de la solidarité et de la cohésion nationale. Or, en moins de trois ans, 7 milliards d'euros ont été économisés par l'État sur le logement des plus défavorisés : ponction budgétaire sur le logement social, baisses des APL, recentrage du au détriment des zones rurales, suppression de l'APL accession. Ces choix politiques ont des effets irrémédiables et installent une crise durable de la construction de logements abordables, de la réhabilitation et de la rénovation urbaines, crise dont, clairement, le pays n'avait pas besoin en ce moment. La situation sociale n'a manifestement pas été suffisamment prise en compte par le Gouvernement dans le plan de déconfinement. Il faut anticiper beaucoup plus et aider les plus fragiles à traverser cette crise. L'urgence est bien d'aider les personnes fragilisées par cette dernière à conserver leur logement. Les aides au logement ont un rôle fondamental. Dans cette période de fragilité pour les Français, elles jouent plus que jamais leur rôle d'amortisseur de la crise. Nous demandons également la suspension de la réforme des modalités de prise en compte des ressources pour le calcul des aides telle qu'elle est envisagée aujourd'hui- sa Alors que les jeunes seront particulièrement touchés par cette réforme, aucune mesure d'accompagnement n'a été prévue par le Gouvernement. Aussi demandons-nous au Gouvernement de revoir les modalités de mise en oeuvre de sa réforme pour mieux accompagner l'installation des jeunes qui entrent dans la vie active.

disons que, collectivement, nous cherchons de l'argent pour financer les APL. Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous vanter- c'est en ce point que, vraiment, je ne comprends plus le discours du Gouvernement -les qualités de votre réforme

Nous aurions souhaité que la trêve hivernale, qui a été prolongée jusqu'au 10 juillet, le soit encore davantage, pour aller jusqu'à l'année blanche totale. Nous avons cependant entendu ce qu'a dit le Gouvernement par la voix du ministre qui était alors chargé de la ville et du logement : il a assuré que « seules les procédures d'expulsion locative adossées à des possibilités de relogement opérationnelles seraient mises en oeuvre à partir de juillet

Notre amendement vise à anticiper les conséquences de la suspension des expulsions locatives pour 2020 en augmentant de 10 millions d'euros supplémentaires l'ouverture de crédits proposée à l'état B dans le projet de loi de finances initiale.

Le budget public consacré à ce projet comprend ainsi, outre 160 millions d'euros de subventions au titre des investissements d'avenir, 123 millions d'euros de crédits budgétaires répartis entre la mission « Culture » et la mission « Recherche et enseignement supérieur Face aux conséquences économiques de la pandémie de covid-19 et devant la dégradation vertigineuse de nos comptes publics, notre estimé et excellent collègue Vincent Delahaye propose, deux amendements, de réduire une partie du financement public du projet par annulation de ces crédits budgétaires. Le présent amendement vise les 97 millions d'euros ouverts au titre du programme « Patrimoines » de la mission « Culture Je vous l'avais dit en ouverture de nos débats : de grâce, discutons des priorités ! Je défendrai tout à l'heure un second amendement, complémentaire de celui-ci, tendant à annuler les 26 millions d'euros de crédits budgétaires imputés sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ». Quel

logique économique qui n'a pas été dévoilée par les auteurs de l'amendement. Le principe est que le Grand Palais réalise une partie des travaux grâce à un emprunt qu'il va

arrivons vraiment aux limites d'un système qui exige des entreprises culturelles qu'elles financent elles-mêmes le remboursement des emprunts qu'elles contractent pour réaliser leurs travaux de rénovation. C'est une absurdité ! Je suis entièrement d'accord avec vous.

Or ce sont ces grandes plateformes qui ont bénéficié de la crise pandémique ; elles n'ont pas besoin d'être renforcées par ce type de produit. Il nous semble beaucoup plus intéressant de mettre à profit les expériences des territoires, parce qu'il se

D'un montant un peu inférieur à ce qui est proposé, ils correspondent à la réalité d'un besoin que nous avons identifié. Surtout, le ministère de la culture a travaillé opérateur par opérateur, en tenant compte aussi du niveau de trésorerie et des disponibilités de chacun.

à des travaux d'analyse du secteur culturel post-crise sanitaire. Les conséquences seront

D'une part, le soutien de l'État à ces opérations crée un effet de levier et entraîne donc plus d'activité et de chiffre d'affaires pour les entreprises, dans la mesure où des subventions des collectivités, des aides d'association et une prise en charge des travaux par les propriétaires privés s'ajoutent aux crédits de l'État.

C'est la raison pour laquelle la commission de la culture plaide pour que ces crédits puissent aussi servir à financer des chantiers d'entretien, dont le lancement est à la fois plus facile et rapide. amendement vise à financer l'action Monuments historiques et patrimoine monumental du programme 175 par un transfert en provenance de l'action Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle du programme 224.

il y manque 100 médecins, et sans les 3000 réservistes qui lui permettent de fonctionner encore, ce service serait en grande difficulté, car il est en tension permanente à cause d'une augmentation massive des interventions.

vous avez noté que la loi de programmation militaire avait prévu l'inversion de la tendance subie par le service depuis plusieurs années. L'objectif du ministère des armées est bien d'aller au bout de cette réforme et de cette montée en charge.

Cet amendement vise à augmenter les effectifs Haut Conseil pour le climat, en les faisant passer de 6 à 24. C'est une modification de crédits modeste, à hauteur de 2,6 millions d'euros, mais qui aura un effet puissant, dont nous avons plus que jamais tenu des enjeux. Cette création permettrait au Haut Conseil pour le climat de mener à bien l'ensemble de ses missions qui, au vu de l'urgence climatique actuelle, sont amenées à croître. En effet, cette instance est un organisme indépendant chargé d'émettre des avis et recommandations précieuses sur la mise en oeuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux, en particulier l'accord de Paris,

en cause, bien sûr, la crise sanitaire, mais pas seulement. Le volume de travail est particulièrement important. Il est impossible, par exemple, d'étudier les hypothèses de la stratégie nationale bas carbone, qui vient d'être publiée, la crédibilité des objectifs de développement de l'hydrogène, ou encore l'incidence de la biodiversité des cibles que la France s'est fixées en matière de méthanisation. La situation n'est pas près de s'arranger, car le Haut Conseil a été invité récemment à étendre encore son champ d'études en y intégrant les problématiques d'adaptation au changement climatique. Pour l'ensemble de ces raisons, et parce que nous considérons que cet organisme est un atout puissant pour les politiques publiques et la transition écologique, nous souhaitons lui donner des moyens suffisants. Quel

donner par avance l'avis du Gouvernement sur les amendements déposés par MM. Longeot, Labbé et Gontard, qui proposent d'abonder le même budget à hauteur de 500 millions d'euros.

l'amendement n° 588 rectifié. Il a déjà été bien défendu, mais j'ajouterai que les acteurs de la filière estiment que, moyennant un renforcement des investissements et des soutiens publics, il est possible et nécessaire de doubler la part modale du fret ferroviaire à l'horizon 2030.

à la congestion des routes, à la pollution de l'air et aux accidents. Il faudrait aussi- c'est une demande sociale forte -, développer les trains de nuit. Une pétition en ce sens a récolté plus de 160 000 signatures. Pour cela, je le répète, il faut massifier les investissements. Le réseau des petites lignes mérite, lui aussi, d'être renforcé. Ces financements sont nécessaires non seulement pour atteindre nos objectifs climatiques, qui font partie de l'urgence, mais aussi pour aménager le territoire de manière équilibrée. Pour combiner relance économique et écologie, cet amendement nous semble

elle ne va pas dans le sens du développement de l'industrie automobile, mais il va falloir faire face à ces paradoxes : le vélo, est-ce de la décroissance ? Non, c'est de la croissance vertueuse ! On doit aller vers la croissance vertueuse et,

qu'elles programment des investissements pérennes en profitant de l'engouement lié à cette crise. l'intérêt du dispositif, vous nous répondez que ce n'est pas le bon moment. Il me semble pourtant, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, que vous n'avez pas pris en compte la nécessité pour les collectivités d'avoir de la visibilité pour planifier ces investissements assez lourds. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

On ne reviendra pas en arrière. Les collectivités doivent donc, dès aujourd'hui, obtenir des moyens de l'État pour transformer ces pistes provisoires en pistes définitives. C'est maintenant qu'il faut le faire : on ne va pas utiliser jusqu'à la fin de l'année les pistes provisoires, qui sont très dangereuses.

au chèque énergie. En effet, depuis la crise, la consommation d'énergie des ménages a véritablement augmenté. En outre, la crise a placé les consommateurs d'énergie face à des difficultés spécifiques. les sénateurs sur ce point, le 21 avril dernier, le médiateur national de l'énergie a déploré l'existence de retards dans les opérations de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, de pratiques de démarchage téléphonique agressives de la part de certains fournisseurs, ou de difficultés dans l'acheminement du chèque énergie. Or la précarité énergétique constitue l'impensé de la gestion de la crise : en effet, la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 n'a prévu pour les ménages qu'un report de la fin de la trêve hivernale ; celui du paiement des factures d'énergie était réservé aux microentreprises. Dans ce contexte, il est nécessaire de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique en revalorisant substantiellement le chèque énergie, dont le montant, établi entre 48 et 277 euros, est bien trop faible pour couvrir les dépenses de consommation d'énergie, mais aussi de rénovation énergétique, auxquelles il donne droit. Quel est l'avis de

au moment de l'achat demeure trop important. Un prêt à taux zéro permettrait de remédier à cette difficulté, car les véhicules non polluants coûtent moins cher à l'usage du fait des économies de carburant réalisées, ce qui permet par la suite le remboursement du prêt.

lorsqu'il s'agissait d'argent public, notamment lors de l'examen des amendements concernant les Français de l'étranger, on savait fixer des critères

Qui gérera quoi ? Vous annoncez que l'Ademe se chargera des projets industriels de décarbonation, l'ASP de l'accélération de l'adoption des technologies de l'industrie du futur-

Essayons de combler le retard en la matière. C'est l'objet de cet amendement que je conçois bien sûr comme un amendement d'appel compte tenu de la règle de recevabilité financière. Toutefois, j'aimerais que le Gouvernement s'engage à combler le retard provoqué par la période de confinement et à accélérer ce plan. C'est sans doute le meilleur moyen d'assurer l'égalité entre territoires ruraux et territoires urbains.

public : créés sur l'initiative des filières industrielles, financés par elles, ils sont des organismes de recherche collective, chargés de faire « ruisseler » l'innovation et la recherche et développement jusqu'aux plus petites entreprises. Ils sont implantés dans les territoires français, sur environ sites au plus près des PME. Nous savons que les mois et années qui s'annoncent se caractériseront par une baisse de l'investissement des entreprises, dont les marges et la trésorerie ont souffert. Les PME seront les plus touchées

entraînant des plans sociaux et la disparition d'entreprises. Il a fallu près de dix ans à la filière pour se reconstruire. Les mesures annoncées dans le cadre du plan Tourisme semblent imparfaites,

-5010Z et 5020Z, qui concernent la location de bateaux avec équipage. Vous avez ajouté la catégorie 7721Z, location et

en direction des CCIFI. Véritable colonne vertébrale de notre dispositif économique à l'export, le réseau des CCIFI a l'habitude de compter sur ses propres forces, en vendant des services et en organisant des événements, puisqu'il ne bénéficie d'aucun financement public. Si nos chambres et leurs membres ne coûtent rien au contribuable, à l'inverse, l'État les sollicite de plus en plus au travers de mécénats pour permettre à la France de tenir son rang à l'international. Aujourd'hui, ce fondé exclusivement sur l'initiative privée conduit certaines de nos chambres à réduire leur budget de fonctionnement. ont déjà suspendu leur activité. Les conséquences de la crise sanitaire justifient d'apporter un soutien ponctuel de 3 millions d'euros au travers de la structure centrale du réseau des CCIFI. Cela permettrait de consolider le réseau mondial de chambres de commerce et d'industrie et de sortir de la crise en ayant la capacité de favoriser la reprise de nouvelles parts de marché, dont nous aurons besoin pour relancer notre économie. C'est urgent ! C'est maintenant ! Cinq suspensions

pour réanimer ce réseau.

et la protection des consommateurs au sein du marché national et européen. Il s'agit donc d'augmenter le budget de la DGCCRF dans l'objectif d'accroître ses effectifs dédiés au contrôle du respect des normes. Cette proposition est issue des travaux de la cellule de veille, de contrôle et d'anticipation « Industrie » de la commission des affaires économiques. Quel Défavorable.

Plus d'un millier de distributeurs de journaux ne recevaient plus ou recevaient très partiellement les quotidiens et les magazines. Cette perturbation résulte de déboires de l'entreprise Presstalis, qui, accablée de dettes, traverse actuellement sa troisième crise majeure en dix ans. Elle a été placée en redressement judiciaire le 15 mai prévoit d'allouer à Presstalis 200 millions d'euros d'aides sous forme de subventions et de prêts du fonds de développement économique et social. Cette aide s'ajoute à l'appui financier important que consent l'État à cette entreprise depuis des années.

du Gouvernement ? Compte tenu du risque systémique que faisait peser une liquidation judiciaire de l'ensemble de la messagerie sur la filière presse,

de tenir compte du risque systémique qui concernerait tout le secteur de la presse. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a pris la décision d'apporter ce soutien en souhaitant que celui-ci permette une véritable restructuration et modernisation de l'opérateur. La parole

Les contenus plus « magazines », la vérification de faits et les enquêtes ont largement favorisé les formats numériques plus réactifs ou les médias nationaux jouissant d'une aura supérieure et d'un accès plus important aux spécialistes. C'est donc tout un modèle éditorial que la presse locale a dû reprendre, et qu'elle va devoir retravailler dans les mois à venir. Cela ne se fera pas sans moyens,

J'espère ainsi que nous pourrons avancer sur cette question.

tonnes de tourteaux de soja- seuls 450 000 d'entre eux sont sans OGM -, lesquels sont utilisés massivement pour nourrir les animaux dans les élevages porcins et bovins. Cette situation est d'autant plus inacceptable

Il y a urgence à relancer la politique de la ville et à impulser une dynamique dans les quartiers. Il faut relancer les opérations de rénovation urbaine, placer l'école au coeur de la politique de la ville, soutenir le tissu associatif. Nous proposons pour cela de créer 30 000 emplois aidés dans les quartiers, afin notamment de mobiliser les jeunes.

s'élevait à 12 000 euros sur trois ans pour les moins de 26 ans, à raison de 4 000 euros par an. C'est vrai qu'il faut éviter des effets de guichet, mais ces dispositifs sont terriblement efficaces.

J'ai rappelé tout à l'heure à M. Savoldelli les dispositifs mis en oeuvre par le Gouvernement pour les ménages les plus modestes. Nous avons clairement préféré affecter les moyens dont nous disposons

les aider à reconstituer leurs droits, il est proposé, à l'instar de ce qui a été fait pour les intermittents du spectacle, de leur accorder une sorte d'année blanche et de créer un revenu de remplacement des CDD d'usage. Le coût d'un tel dispositif s'élèverait à

les discussions sur le soutien à tel ou tel secteur économique. Je le regrette très profondément, parce que je crois que nous ne prenons pas la mesure de la situation. situation. Cet amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 50 millions d'euros en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à la gestion de l'épidémie de covid-19.

Je déplore que ces différentes propositions ne soient pas adoptées, que nous ne prenions finalement jamais le temps de vraiment débattre et de montrer aux Françaises et aux Français que nous avons conscience de la situation sociale dans laquelle nombre d'entre eux se trouvent.

Ce sont des amendements miroirs avec ceux qui ont été examinés en première partie. Il s'agit non pas d'une prime pour les salariés des Ehpad, mais d'une demande de financement de prime pour les salariés des sous-traitants dans les Ehpad. Nous avons indiqué en première partie que les sous-traitants

Cet amendement vise à ouvrir 120 millions d'euros de crédits, afin de nationaliser les sociétés Luxfer, Famar et Péters Surgical. Pour rappel, la seule réponse à la pénurie de masques de protection et de tests de dépistage que nous avons connue lors de la pandémie a été un rationnement de leur utilisation, sans entrer plus avant dans la polémique. Après cette pénurie de masques, de tests de dépistage, de médicaments il y a quelques mois, nous ne pouvons que constater que la France est totalement dépendante et extrêmement fragilisée sur le plan sanitaire. Pourtant, des entreprises sur le territoire français ont encore un savoir-faire industriel et pourraient contribuer à inverser la tendance. Trois entreprises en particulier ont besoin de l'intervention de la puissance publique pour continuer à produire. L'entreprise Luxfer, à Gerzat, était jusqu'en 2019 la seule en Europe à fabriquer des bouteilles d'oxygène à usage médical. La société Famar, spécialisée dans la production de chloroquine, est actuellement en redressement judiciaire. l'entreprise Péters Surgical à Bobigny, conceptrice des sondes de Montin utilisées en réanimation est menacée d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ces trois entreprises sont indéniablement des secteurs stratégiques,

cela peut concerner des clusters tel celui de Magny-Cours dans la Nièvre, où 39 entreprises interviennent dans les domaines de la haute technologie, de l'industrie automobile du sport de compétition et de loisir, de l'aéronautique et de la R&D relative à la voiture de

Catherine Conconne. Il s'agit de créer une prime pour le climat et l'élimination des passoires thermiques. On parle d'écologie, de lutte contre le réchauffement climatique, mais pour l'instant tout cela reste très théorique, avec des hauts conseils, des bas conseils, des moyens conseils ... Nous avons l'occasion d'entrer dans du concret.

Le transport public français se trouve dans une situation grave du fait des baisses de versement mobilité.

Nous nous félicitons de la création d'un ministère dédié à la mer. Cependant le secteur portuaire reste un grand absent de ces plans de relance, alors qu'il joue un rôle central en matière d'aménagement du territoire et de transition écologique. Le rapport de la mission d'information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes, dont Michel Vaspart était le rapporteur et Martine Filleul la présidente, a été présenté le 1 juillet dernier. Il estime nécessaire un véritable plan de relance, sans attendre

pour les collectivités locales, à hauteur de 500 millions d'euros en crédits de paiement pour l'année 2020.